La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

si l'on peut dire, les obligations de construction dans les villes carencées au regard de la loi SRU. Actuellement, dans ces villes, toute nouvelle opération de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface habitable doit comprendre au moins 30 % de logements sociaux.

nous estimons qu'il convient de replacer les obligations de mixité sociale au rang d'alpha et d'oméga de toute opération de construction, lorsqu'il s'agit de villes carencées. Peut-être ces opérations n'intéressent-elles pas les bailleurs, mais c'est le sens de l'histoire que d'aller vers une meilleure mixité sociale, à une échelle toujours plus petite, de la ville au palier. D'ailleurs, il n'est pas utile de se faire des noeuds au cerveau : si c'est là la seule manière de construire, et si la ville est dotée d'un office public de l'habitat, alors cet office, sur demande de la collectivité, pourra à l'évidence prendre en charge la gestion et le coût de cette construction. Lorsqu'il Lorsqu'il existe une volonté, il y a toujours une solution. D'ailleurs, nous le voyons bien, cet exemple illustre la nécessité de disposer d'organismes d'HLM à taille humaine, en capacité de faire ce travail de « dentellière urbaine Dans le même esprit, nous avions proposé, là où les enjeux de construction de « la ville sur la ville » sont les plus forts, d'appliquer cette règle de 30 % de logements sociaux par opération

Le nombre de logements sociaux à construire reste exactement le même. En revanche, l'adoption de cet article permettrait aux opérateurs de reporter cette création sur une opération voisine, afin de mutualiser les coûts particuliers de conception et de réalisation. Cette disposition nous a semblé de nature à encourager la construction de logements. Par ailleurs, il est plus facile, pour les bailleurs sociaux, de gérer un parc de plusieurs dizaines ou centaines de logements sociaux regroupés

à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet dispose de la faculté, et non de l'obligation, de prendre un arrêté de carence de la commune après consultation du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Près d'un tiers des 1 022 communes concernées par le bilan triennal 2011-2013 n'ont pas respecté leur objectif. Or, grâce au pouvoir d'appréciation du préfet, seules 218 communes ont fait l'objet d'un constat de carence, entraînant une majoration de prélèvement. du dernier rapport triennal, sur les 1 152 communes concernées, la moitié n'ont pas respecté leur engagement, mais seules 233 ont été déclarées en situation de carence, soit 36 % des communes concernées, si bien que la commission nationale SRU a demandé et obtenu un relèvement du nombre des communes dont Nous considérons, pour notre part, que l'ensemble des collectivités ne respectant pas leurs engagements triennaux doivent être soumises à une majoration de prélèvement ; les circonstances locales doivent être prises en compte, mais seulement pour la définition du montant de cette majoration -c'est d'ailleurs le cas, puisque la majoration du prélèvement demeure très variable en fonction des circonstances locales et des préfets de région, selon un rapport de l'Assemblée nationale. Il s'agit de mettre concrètement en oeuvre le principe d'égalité des collectivités

902 rectifié , la commission nationale SRU a déjà du mal à faire face aux missions qui lui sont aujourd'hui dévolues ; lui en confier de nouvelles missions,

n° 666 rectifié . Monsieur le ministre, peut-être avons-nous une divergence d'appréciation sur l'alinéa 9 de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'une commune fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l'offre de logement intermédiaire prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d'effet.

Pourtant- et c'est paradoxal, nous en avons parlé tout à l'heure -, le nombre de communes qui persistent à ne pas contribuer à cet effort national de solidarité a augmenté. Des sanctions sont prévues à l'encontre des communes qui ne respectent pas leur obligation ; visiblement, il faut encore les renforcer.

avis défavorable sur cet amendement. Les opérations de transformation de bâtiments existants sont très coûteuses. Imposer des obligations très contraignantes de production de logement social fragiliserait l'équilibre financier

Ce projet contient donc intrinsèquement les germes de nouvelles ségrégations urbaines et sociales. Or nous estimons qu'il est du ressort du législateur de définir les règles communes qui permettront d'éviter ces écueils et de soumettre ce développement urbain à l'intérêt général. Notre proposition est simple. Il s'agit d'affirmer que, dans toute construction nouvelle de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface habitable et située à moins de 400 mètres d'une nouvelle gare, la proportion de logements locatifs sociaux devra être, au minimum, de 30 %. Il ne s'agit pas de chambouler les normes existantes, puisque cet objectif de 30 % de logements sociaux est déjà inscrit dans le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF, approuvé à la fois par l'État et par la région.

Dans ces villes-là, la proportion de logements sociaux diminuera donc mécaniquement. Il importe que nos villes restent des villes populaires et que l'arrivée du métro ne conduise pas à l'éloignement du centre des habitants modestes.

de la loi sur le Grand Paris impose aux contrats de développement territoriaux d'établir des diagnostics en matière de logement, puis de préciser le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser au sein des périmètres concernés. L'article 24 de cette même loi dispose que, dans les communes concernées par la loi SRU, les actions ou opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures prévus autour des gares du Grand Paris

peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, demander au propriétaire le loyer de référence de l'appartement. Le présent article prévoit la suppression de cette possibilité. Nous pensons que la connaissance du loyer de référence est importante pour que le locataire puisse estimer si le montant de son loyer est raisonnable. Après l'abandon de l'encadrement des loyers, on supprime ici un droit du locataire : celui d'estimer lui-même si son loyer est trop élevé ou non. Quand on fait des lois sur la confiance,

Quel est l'avis du Gouvernement ? à rétablir dans le contrat de location la mention relative aux loyers de référence qui sont établis pour la mise en oeuvre de l'encadrement du niveau des loyers. tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit la mention des loyers de référence dans les contrats de location signés pour les logements situés dans les zones où s'applique l'encadrement du niveau des loyers. Le dispositif d'encadrement du niveau des loyers étant transformé en dispositif expérimental au travers de l'article 49 du projet de loi ÉLAN, il convient d'en tirer les conséquences dans la loi de juillet 1989. Cette mention, très logiquement, ne sera insérée dans le contrat de bail que dans la mesure où le logement se trouvera dans une zone où l'encadrement des loyers sera effectivement expérimenté, en application de l'article 49 du projet de loi. C'est la raison pour laquelle la disposition ne

Cet amendement vise à préciser que les associations représentatives des locataires peuvent figurer dans la liste des personnalités qualifiées. Disposant d'un savoir-faire et d'une expertise acquise sur le terrain et dans les conseils d'administration des organismes d'HLM, les associations représentatives peuvent à ce titre être désignées comme personnalités qualifiées. Les associations représentatives des locataires sont en effet des acteurs incontournables du logement. Premiers interlocuteurs entre locataires et bailleurs, organisées au plus près des locataires, elles assurent quasiment une mission de service public et sont subventionnées pour leur utilité sociale et leur mission d'intérêt général.

À l'initiative d'avancées significatives et de projets qui mettent au coeur le vivre ensemble, comme l'emblématique fête des voisins ou de nombreuses mobilisations citoyennes, ces associations ont toute leur place au sein des observatoires locaux des loyers. Ainsi, au vu de l'action et de l'implantation des associations représentatives des locataires dans le paysage français, il convient de les désigner comme personnalités qualifiées afin qu'elles puissent participer aux organes dirigeants des observatoires locaux des loyers. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

Si nous défendons l'encadrement des loyers dans son principe, c'est son application selon l'article 49 que nous condamnons. L'encadrement des loyers prévu par le projet de loi D'une part, étant optionnel et temporaire, il enterre les caractères d'automaticité et de durabilité du dispositif ALUR de 2014. Le caractère « expérimental » de l'encadrement des loyers semble particulièrement superflu, dans la mesure où le dispositif ALUR, qui a été en vigueur pendant près de quatre ans à Paris et à Lille, a déjà montré des effets positifs en termes de stabilisation des prix. L'augmentation des loyers est passée de 10 % avant 2015 à seulement 1 % après la mise en place de l'encadrement. À Paris, dès le lendemain de la décision du tribunal administratif de supprimer le dispositif, certaines annonces des sites de location affichaient des loyers supérieurs de 30 % à ceux D'autre part, l'ambiguïté juridique autour des critères et conditions- « un écart important entre le niveau de loyer moyen du parc privé et du parc social » ou encore « un niveau de loyer médian élevé

le pouvoir décisionnel et appréciatif concernant les critères, laissant à la collectivité un simple pouvoir de négociation. À cela s'ajoute la complexité juridique de cette politique, que l'on retrouvait aussi dans la loi ALUR de 2014. La décision du Conseil d'État du 15 mars 2017 d'annuler l'encadrement des loyers, restreint par le gouvernement Valls à Paris et à Lille, a mis en cause non seulement la faiblesse du périmètre d'application, mais aussi la complexité du dispositif ALUR, par lequel la loi s'applique après prise d'un décret d'application puis d'un arrêté par chaque préfet. Si « simplification » semble être le mot d'ordre du Gouvernement, désireux de casser les acquis collectifs de notre République, il semble lui préférer la complexification juridique lorsqu'il s'agit de réguler le marché. Pourtant, une régulation des loyers obligatoire dans toutes les communes dites « tendues » et mise en place par la loi permettrait le contournement des problèmes que pose l'insécurité juridique et garantirait efficacité et pérennité dans l'encadrement des loyers, cela dans le respect du principe d'égalité territoriale.

l'amendement n° 222. Nous ne souhaitons pas que l'encadrement des loyers devienne une simple expérimentation fondée sur le volontariat des collectivités, car cela risque encore de creuser les inégalités entre nos concitoyens selon leur lieu de résidence. Encore une fois, le dispositif d'encadrement n'a nullement été censuré sur le fond. L'expérimentation que vous nous proposez revient, au final, à ne pas choisir et à se défausser sur les EPCI ou sur les autorités compétentes en matière de logement. Pourtant, la crise du logement en zones tendues n'est plus à démontrer. Les gens sont étouffés par des loyers exorbitants, justifiés par la seule spéculation, par le seul appât du gain. On nous parle de pénurie de logements, d'écoeurement des spéculateurs, de refus de prendre des risques, de crise de l'immobilier on croit rêver ! À Paris, par exemple, 40 % des logements loués le sont à un prix supérieur au maximum autorisé par la réglementation. La pression sur les ménages est toujours plus forte et personne n'est épargné. Il est hallucinant de voir comment les intérêts d'une minorité des fonds de pension, de surcroît, priment encore une fois l'intérêt général, l'intérêt de nos concitoyens ! Il est du devoir de l'État d'intervenir et de juguler la rente de l'immobilier, qui se développe. L'État doit s'impliquer et jouer son rôle de régulateur. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. L'amendement n° 1054 rectifié n'est pas soutenu. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 222 ?

Le dispositif d'encadrement des loyers tel qu'il est prévu dans la loi ALUR n'est pas sécurisé. On me répondra que c'est une question de forme, pas de fond. Il n'en reste pas moins qu'il a été

pris la décision de saisir le Conseil d'État pour être cohérent et logique avec la position que m'avaient demandé d'adopter la maire de Lille et celle de Paris.

Il est précisé que l'encadrement des loyers peut s'appliquer sur une partie seulement du territoire de l'intercommunalité, en réponse aux décisions d'annulation des tribunaux administratifs de Lille et de Paris. Entré en vigueur le 1 août 2015 à Paris et le 1 février 2017 à Lille, l'encadrement des loyers a fait ses preuves. Sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, on constate une quasi-stagnation des loyers entre 2016 et 2017, qui contraste fortement avec des hausses annuelles voisines de 6 % de 2006 à 2013. Par ailleurs, le dispositif est, depuis l'origine, mesuré. Il vise surtout à bloquer les loyers abusifs, au-delà de 20 % d'un loyer de référence fixé selon les prix du marché.

à nouveau par voie d'expérimentation. L'amendement vise donc à pérenniser ce dispositif pour assurer une meilleure visibilité de la mesure aux villes qui souhaitent le mettre en place. Quel est l'avis de la commission ? Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement

L'article 49 tend à tirer les enseignements des difficultés rencontrées dans l'application du dispositif d'encadrement du niveau des loyers depuis 2014. À ce titre, le dispositif est tout d'abord rendu optionnel et expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Les expérimentations menées dans plusieurs grandes villes de France ont produit des résultats probants, permettant la sécurisation des bailleurs et des locataires dans le parc privé.

deux ans pour demander à appliquer le dispositif d'encadrement des loyers. En commission, nous nous sommes déjà prononcés sur l'amendement de M. Bargeton. Nous avions donné un avis favorable, sous réserve qu'il soit rectifié pour réduire le délai à un an.

fallait des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le PLH, ainsi que de faibles perspectives d'évolution de celui-ci. D'un point de vue juridique, qu'appelle-t-on un taux de logements commencés faible par rapport, par exemple, au nombre de logements à Paris ? à Paris ? C'est assez difficile à définir. Par ailleurs, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter ces deux critères, sauf à penser que le taux de construction est si important qu'il serait de nature à réguler les prix.

une régulation des prix ? J'en doute. Indépendamment de ce doute, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter ces deux critères, qui me paraissent inutiles. Je propose donc que nous supprimions ces deux alinéas.

Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont : lors de la préparation du texte, le Conseil d'État nous a expliqué que ces critères étaient tout à fait utiles, et même indispensables. Il nous arrive de suivre les avis du Conseil d'État

Les bailleurs sociaux voient déjà leurs loyers fortement encadrés, au niveau tant des plafonds que des loyers pratiqués. Le loyer maximum des nouvelles conventions est fixé chaque année, par circulaire, en janvier. L'autorité administrative fixe pour les loyers un montant minimum et un montant maximum, établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge des organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien. Dans les deux cas, les loyers fixés ne pourront être révisés chaque année à la hausse, au 1 janvier, que dans la limite de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre. Ajouter un nouveau cadre à celui-ci ne nous paraît pas judicieux. Cet amendement tend à préciser que tel ne sera pas le cas.

majoré sur la base d'un indice clair, précis et fiable, celui du montant du loyer plafond du prêt locatif social fixé par l'État. Nous préconisons donc que le loyer de référence soit défini par rapport au plafond de loyer pour les logements financés par le dispositif du prêt locatif social, le PLS, qui, tout en étant du logement social, se situent dans une fourchette particulièrement élevée. La référence du PLS permet de fixer avec précision le loyer de référence, puisqu'il s'agit d'un indice fixé chaque année par le représentant de l'État. De plus, une telle intégration se justifie pleinement, pleinement, nombre de personnes relevant du logement social se logeant aujourd'hui dans le privé, faute d'une offre adaptée. Autre avantage à nos yeux, un tel mécanisme de fixation du loyer médian de référence, en le déconnectant de l'existant, permet de faire baisser instantanément les prix du loyer.

Quel est l'avis du Gouvernement ? L'amendement vise à prévoir que le loyer de référence majoré est fixé administrativement au niveau du loyer maximum du prêt locatif social applicable aux logements sociaux. la fixation du loyer de référence majoré, qui est le résultat des observations de l'observatoire local des loyers du territoire concerné, est le reflet du marché locatif. Le projet de loi qui est soumis à l'examen de la Haute Assemblée n'a pas changé cette modalité de fixation du loyer de référence. Il ne me semble pas opportun d'en modifier les modalités de fixation. Une évaluation du dispositif expérimental permettra d'en tirer toutes les conséquences et de proposer, le cas échéant, des modifications.

: La parole est à M. Guillaume Gontard. L'article 50 supprime l'adaptation des règles de décence dans les hôtels meublés, sous couvert de la difficulté d'édicter un corpus minimal de règles, mais surtout pour éviter le coût financier de l'adaptation des locaux. Pour rappel, quelque 25 000 personnes en grande urgence sociale sont actuellement logées dans ce type de logement. Encore une fois, ce projet de loi est l'inverse de ce qu'il affiche ; il ne lutte pas contre ce qu'il prétend combattre. Vous renoncez purement et simplement aux ambitions qui devraient tous nous animer l'édiction de véritables règles de décence pour l'hébergement des plus démunis, alors même que celui-ci constitue bien souvent le premier facteur de dignité. Vous proposez tout de même que l'on se passe d'un article du code de la santé publique Par ailleurs, en cas de colocation à baux multiples, le projet de loi prévoit que les conditions de décence soient appréciées en prenant en compte l'ensemble des équipements, éléments et pièces du logement. C'est faire peu de cas de la réalité. Il n'est pas question pour nous de viser la colocation étudiante- et quand bien même ! -, mais le fléau des marchands de sommeil. Par exemple, la division de pavillons en chambres de 9 mètres carrés pourra « aboutir à la coexistence d'autant de ménages, au partage d'équipements insuffisants pour leur nombre- toilettes, salle de bains -et à une dégradation rapide du bien et des conditions de vie de ses occupants », soulignait la Fondation Abbé Pierre. Comble de tout, vous consacrez un seul article à ces enjeux majeurs pour certains territoires ! Devons-nous rappeler, encore une fois, le chiffre inacceptable du développement du logement insalubre ? Celui-ci représente 40 % des logements dans certaines villes autour de Paris, où la responsabilité de l'État est engagée pour une large part. Les élus locaux pointent la difficulté logistique de la lutte contre les marchands de sommeil. La justice possède peu de moyens face à la rapidité de tels délinquants. J'ai peur qu'ils en aient encore moins Nous appelons vivement nos collègues à voter la suppression de cet article, qui consacre l'indignité et laisse le champ libre aux marchands de sommeil.

L'amendement a pour objet de supprimer l'article relatif à l'application des règles de décence aux colocations et aux hôtels meublés loués en tant que résidence principale. bien clair, que la volonté du Gouvernement est non pas de créer de nouvelles règles de décence pour des locaux loués à usage de résidence principale dans les hôtels meublés ou dans les colocations, mais bien d'appliquer les mêmes règles pour tous. règles pour tous. S'agissant plus particulièrement des hôtels meublés, ceux-ci ne sont pas destinés à constituer des logements pérennes. Ils assurent l'hébergement de personnes sans domicile, avant que ces dernières puissent être relogées, même si l'expérience a montré qu'elles peuvent y résider plusieurs années. Néanmoins, lorsque ces locaux deviennent des logements, les personnes qui y résident bénéficient des règles de la décence, et il faut qu'ils en bénéficient. peut imposer le respect de ces règles de décence s'il est amené à requalifier le contrat d'occupation en contrat de location. Il n'est donc pas utile de prévoir des règles spécifiques de décence pour l'occupation. Si vous supprimez cet article, l'amendement aura un effet strictement contraire à ce que vous souhaitez, puisque ne sera plus permise l'application des règles générales de décence inscrites dans la loi de 1989 aux hôtels meublés.

collaboratives. La loi permet évidemment aux services municipaux ou départementaux du logement d'accéder à ces locaux, mais elle ne prévoit pas l'obligation d'accéder aux parties communes.

Afin de rendre conformes les règles de la copropriété, il faut indiquer dans la loi que le syndic désigné de l'immeuble doit permettre aux agents du service municipal du logement qui en feraient la demande d'accéder aux immeubles

concernés. Quel est l'avis de la commission ?

Renforcement de la spéculation immobilière, renchérissement des prix, aggravation de la pénurie de logements accessibles entraînant une baisse du nombre d'habitants dans les coeurs de ville, nuisances de voisinage, détérioration du tissu commercial et de la vie de quartier comme l'a récemment détaillé la mairie de Paris par voie de communiqué, les plateformes de location meublée de courte durée- on pense notamment à Airbnb, mais ce n'est pas la seule -ne sont pas uniquement une source de jouissance pour les locataires qui en bénéficient et pour les loueurs qui en profitent ... Et pour cause ! Le Le développement de ces locations de courte durée peut notamment entraîner des troubles de voisinage englobant nuisances sonores, dégradation des parties communes, etc. Une tentative de résorption du phénomène avait été enclenchée avec la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme qui prévoyait initialement l'obligation pour un copropriétaire de saisir l'assemblée générale pour toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation, aux fins de location pour des courtes durées à une clientèle de passage. Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2014-691, que cette disposition portait une atteinte disproportionnée aux droits des copropriétaires ; il l'a, de ce fait, censurée. Nous proposons, au travers de cet amendement, un autre moyen de contraindre les bailleurs, en permettant aux copropriétaires de modifier le règlement de copropriété et en assouplissant les règles de majorité, afin d'interdire l'exercice de toute activité professionnelle ou commerciale dans les lots d'habitation. Il est évident qu'en conservant la règle de l'unanimité, nous ne pourrons résoudre ces problèmes. Le plus souvent, il s'agit d'une majorité de propriétaires qui vivent dans leurs logements et d'un ou deux locataires qui créent des nuisances dans l'immeuble. Les gens ne peuvent plus dormir, et les parties communes sont souvent souillées par des locataires qui se sentent peu concernés par les règles de vivre ensemble au quotidien. Cette disposition ne pourra aucunement être qualifiée d'excessive puisqu'elle contraindra seuls copropriétaires louant leur logement pour plus de cent vingt jours par an à une clientèle de passage, la location pour une durée inférieure n'étant pas affectée par une telle clause. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à protéger l'ensemble des habitants d'un même immeuble subissant les nuisances de certains occupants de courte durée, irrespectueux de la vie en communauté. Quel est l'avis de la commission ?

Nous abordons, avec cet article, le sujet du développement des plateformes de location de biens immobiliers pour de courtes durées, c'est-à-dire Airbnb et ses équivalents. le développement de ces plateformes pose une série de difficultés aux collectivités concernées et à leurs habitants. Premièrement, en dehors des cas de sous-location de chambres ou de location de courte durée du logement principal, cette pratique a pour conséquence directe de soustraire au marché locatif un nombre croissant de logements. Elle participe aussi à la hausse des prix du marché immobilier en accroissant le déficit de l'offre par rapport à la demande. On assiste ainsi à un phénomène de désertification des centres-villes, des habitants étant chassés vers la périphérie pour accueillir les touristes aisés ou la bourgeoisie mondiale de passage. Par ailleurs, beaucoup d'acteurs du tourisme considèrent que ces plateformes font une concurrence déloyale au secteur hôtelier traditionnel, lequel est astreint à une réglementation plus exigeante. Aujourd'hui, très concrètement, du fait de ces pratiques, quelque 26 % des logements sont soustraits du marché locatif dans les quatre premiers arrondissements de Paris. Les autorités locales considèrent que 20 000 logements ont été perdus pour la location traditionnelle en cinq ans. Il y a donc urgence à répondre à ces enjeux. Pour cette raison, nous avons déposé, au mois de mars dernier, une proposition de loi visant à encadrer ces pratiques,

Nous sommes satisfaits de voir que le Gouvernement a fait le choix de s'emparer de ce sujet. Car, loin de l'image d'une économie collaborative, le développement de ce type de pratiques correspond en réalité à une énième dérégulation du marché. Ces plateformes sont en effet de plus en plus utilisées par des professionnels multipropriétaires comme solution de rechange à la location traditionnelle. Il est ainsi bien plus rentable et moins contraignant de faire de la location de courte durée de tourisme, plutôt que de la location traditionnelle, avec les exigences de respect du bail et des droits des locataires Une telle démarche, à la différence de la location de chambres par des particuliers pour de courtes durées, accroît le déficit de l'offre de logements locatifs en zone tendue. Ce n'est pas acceptable puisque, dans ce cas, le développement de l'offre de logements touristiques s'oppose très directement au droit au logement des habitants des métropoles. Nous ferons donc, au travers de nos amendements, des propositions constructives pour renforcer les dispositions du présent article et porter plus loin l'encadrement préconisé.

L'article 51 vient compléter la loi ALUR, qui a instauré le changement d'usage pour les hébergements touristiques et la loi pour une République numérique, qui a ajouté à cette mesure une déclaration préalable soumise à enregistrement dans les zones tendues,

Nous y considérons que le développement de l'offre de meublés de tourisme, qu'il s'agisse de logements dédiés ou de résidences principales, est bienvenu. En effet, il renforce l'activité touristique de notre pays

des spéculateurs multipropriétaires se sont engouffrés dans cette activité de location touristique plus lucrative, et ont ainsi soustrait des logements à la location annuelle en zones tendues. Nous sommes donc globalement favorables à cet article, qui clarifie le cadre de la location meublée touristique

qui donne les moyens aux communes de réguler de façon efficace et crédible l'offre de meublés touristiques, là où il existe une tension sur le marché du logement. L'article ménage un équilibre qui est satisfaisant, comme l'a souligné M. le secrétaire d'État. Les personnes ont

L'objet de cet amendement est de rétablir l'exemption d'obligation de déclaration préalable pour les propriétaires de résidences principales, à l'exception des loueurs utilisant une plateforme numérique non transactionnelle prêtant gratuitement son concours à la mise en location de locaux meublés. Une telle disposition permettrait d'épargner aux hébergeurs consciencieux une contrainte administrative qui avait disparu. À ce stade, il apparaît en effet nécessaire d'éviter d'empiler de nouvelles dispositions sur les mesures existantes. La France est en train de devenir le pays le plus compliqué pour la location meublée, alors qu'elle souhaite demeurer le premier pays touristique et manque d'hébergements dans ce secteur. une telle disposition contribuerait à encourager les loueurs à se détourner de l'économie grise, qui se développe dans le secteur de la location meublée, à la faveur du développement de la réglementation dans ce secteur. En outre, l'obligation de déclaration préalable comme moyen de contrôle est inutile pour les villes. En effet, au 1 janvier 2019, les plateformes de location de vacances en ligne qui réalisent les transactions entre les hébergeurs et les touristes auront l'obligation de collecter automatiquement la taxe de séjour auprès de leurs utilisateurs sur tout le territoire pour la reverser aux communes et communautés de communes. À cette date, la seule taxe de séjour qui leur échappera sera celle qui est liée aux transactions réalisées hors ligne sur les plateformes de mise en relation qui n'assurent pas de service de télépaiement. Il est donc nécessaire de cibler la surveillance sur ce type de plateformes.

en raison du gain de pouvoir d'achat qu'elle peut représenter. Par ailleurs, une telle mesure dénature l'accord équilibré, trouvé en juin dernier entre les plateformes et le Gouvernement, qui comporte des engagements concrets et précis du secteur destinés à répondre aux préoccupations légitimes des villes et des utilisateurs de ces plateformes.

effet, cette déclaration peut être utile, d'une part, pour mieux percevoir la taxe de séjour, notamment dans le cas de location des plateformes non transactionnelles, et, d'autre part, pour permettre aux communes de mener une politique de qualité sur ce type d'hébergement. L'amendement n° 758 rectifié est néanmoins intéressant, car il tend la déclaration simple en mairie lorsque la location est effectuée au travers d'une plateforme non transactionnelle. Pour autant, comme il revient sur la position et l'ajout de la commission,

Viviane Artigalas, pour explication de vote. fasse l'objet d'une simple déclaration en mairie. Ces amendements en discussion commune tendent à revenir sur cette mesure. Ce n'est pourtant pas grand-chose que de demander aux propriétaires de remplir un formulaire avant de mettre leur bien en location. Ce dispositif est, au contraire, utile pour les maires, qui pourront mieux connaître leur parc de meublés de tourisme, quand bien même celui-ci est mouvant, et ainsi mener une politique de qualité dans ce domaine. Il ne s'agit nullement de lutter contre les meublés de tourisme, car je considère que leur développement est un atout pour l'attractivité

car, si les plateformes transactionnelles sont obligées de la percevoir dès 2019, ce n'est pas le cas des plateformes non transactionnelles. On entend dire que la législation en la matière est mouvante et trop lourde, mais quel a été l'objectif du législateur ces dernières années ? Faire en sorte que les revenus perçus soient fiscalisés, comme tous les autres ; faire en sorte que la taxe de séjour puisse être recouvrée ; faire en sorte d'éviter que des biens ne soient soustraits du marché locatif traditionnel et, ici, faire en sorte que le propriétaire ait conscience que louer son bien n'est pas un acte anodin et permettre aux maires d'être mieux outillés pour mener une politique touristique. Sont-ce là des objectifs blâmables ? Des dispositions disproportionnées ? Il ne nous semble pas ! Il s'agit seulement de faire rentrer dans le droit commun des activités qui ont pu se développer à sa marge, et en aucun cas de lutter contre leur développement qui, je le répète, est nécessaire pour répondre aux attentes des touristes.

un certain nombre d'années, nous avons mis, notamment à la commission des finances, tous les sujets liés à l'économie numérique sur la table. Nous avons tout d'abord examiné ce qui touchait à la fiscalité- c'est bien normal à la commission des finances ! -, que ce soit la perception de la TVA sur le e-commerce, mais aussi la fiscalisation

que les choses aient évolué dans le bon sens, car je me souviens de ce que l'on entendait au début. Les plateformes- je ne citerai pas de nom -hurlaient à la mort en disant qu'on allait tuer leur modèle économique ; j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, dans ce domaine

le problème vient, je le crois, de la massification du tourisme partout à travers le monde. Des touristes, il y en a de plus en plus, notamment dans les très grandes villes.

de simplifications, notamment pour les résidences principales. Toutefois, vu l'avis des deux camps, je retire mon amendement,

Nous proposons donc de passer de 120 à 90 le nombre maximal de nuitées autorisées annuellement pour les propriétaires louant leur résidence comme meublé de tourisme les plateformes de réservation, type Airbnb. Ce seuil de 120 jours applicable aux communes ayant adopté le changement d'usage, soit les communes de plus de 200 000 habitants, découle directement de la définition de la résidence principale explicitée par l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Or cet article est antérieur à l'arrivée des plateformes collaboratives, phénomène qu'il n'a par conséquent pas anticipé. Son objet n'a jamais été de constituer un cadre de réglementation pour les locations saisonnières. Il semble nécessaire à nos yeux de revoir le seuil des 120 jours, actuellement trop permissif au vu du contexte global, avec les phénomènes de forte ubérisation du marché immobilier, de concurrence déloyale auprès des hôteliers traditionnels et de tensions en matière de logement. Abaisser le seuil à 90 jours permettra de limiter les conséquences néfastes des locations saisonnières sur les locations traditionnelles, mais aussi d'effectuer une harmonisation avec les visas touristiques de l'espace Schengen, qui sont d'une durée similaire. J'ajoute qu'une limite de 90 jours n'est en aucun cas trop stricte. D'ailleurs, de nombreuses villes internationales ont adopté des mesures bien plus contraignantes, notamment à Amsterdam et San Francisco, où le nombre maximal de nuitées est de 60 jours par an.

Nous ne pouvons pas ignorer que, avec 120 jours, nous sommes dans la fourchette haute des réglementations existant en Europe et en Amérique du Nord, notamment. Nous proposons donc 90 jours. D'ailleurs, quelque 90 % des loueurs sont aujourd'hui en dessous des 120 jours par an. 120 jours par an. Le nombre de nuitées que nous proposons est adapté et vise principalement les multipropriétaires qui cherchent à se spécialiser de manière industrielle dans la location saisonnière. Quel est l'avis de la commission ?

résidences secondaires, sans qu'aucune autorisation soit nécessaire en deçà de ce seuil. À Paris, il n'est pas possible de louer sa résidence secondaire, ne serait-ce qu'une journée, sans autorisation de changement d'usage, donc sans compensation. Le régime en vigueur est donc déjà particulièrement strict. Il nous a semblé disproportionné de devoir le renforcer, et probablement non conforme au droit européen. Nous avons préféré opter pour un système qui maintient un équilibre satisfaisant

pour explication de vote. En l'occurrence, c'est un sujet qui est devant nous, devant l'Europe. Il n'y a pas un droit européen qui nous tombe dessus ! La France doit être à la pointe des pays qui portent ce débat au plan européen avec les grandes villes qui sont concernées, les autres grandes villes françaises. Nous avons un devoir d'anticipation et de création du droit européen, nous ne sommes pas là pour faire comme s'il tombait du ciel. Par ailleurs,

parfois un peu naïve, comme si nous avions face à nous des personnes avec lesquelles nous allions pouvoir discuter facilement. Mais ces plateformes sont des multinationales, qui ont une force de développement importante. D'ailleurs, le phénomène a été extrêmement rapide, et il peut encore s'étendre. Si nous n'envoyons pas un signal législatif fort, nous serons demain, à la faveur des événements internationaux qui vont se tenir en France par exemple, facilement débordés par la croissance de ce phénomène. Il nous faut donc un arsenal législatif dissuasif,

L'article 51 prévoit de recourir au régime d'amende civile, dont le montant peut aller jusqu'à 5 000 euros, y compris pour le défaut de déclaration simple en mairie. cela créerait une différence de traitement difficilement justifiable entre l'absence de déclaration d'une chambre d'hôte et l'absence de déclaration d'un meublé de tourisme, actuellement soumises à la même contravention de 450 euros. C'est pourquoi il est proposé d'en rester au droit en vigueur en ce qui concerne la sanction de l'absence de déclaration simple, à savoir une contravention. En revanche, là où un régime de changement d'usage et une déclaration soumise à enregistrement sont en vigueur, le régime de l'amende civile a toujours vocation à s'appliquer. Cet amendement ne tend pas à revenir

proposons, au-delà de l'amende créée par ce texte, de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour et par annonce pour compléter l'arsenal législatif. Il s'agit ainsi de faire encore plus pression sur les plateformes ne retirant pas les annonces qui ne disposent pas d'un numéro d'enregistrement ou dont la durée légale maximale de mise en location est dépassée. La mise en oeuvre d'une astreinte nous semble ainsi un bon moyen d'atteindre l'objectif visé par cet article le respect de la loi par les plateformes de type Airbnb. Ainsi, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l'annonce, le président du tribunal peut ordonner la suppression de l'annonce dans un délai qu'il fixe. À l'expiration de celui-ci, le juge pourra prononcer

cet amendement. La création du bail mobilité permet de mobiliser un parc de logements qui n'auraient pas été loués sans ce nouvel outil, notamment dans les métropoles et villes étudiantes où le le besoin de baux de courte et moyenne durées est important. En incitant les propriétaires à avoir

l'article 34, qui instaure le bail mobilité, améliore déjà substantiellement la situation des propriétaires de pied-à-terre, en leur permettant de louer leur résidence secondaire en bail mobilité

en renvoyant expressément au décret fixant la liste des communes pour lesquelles une autorisation de changement d'usage peut être instaurée par celles qui le souhaitent. À l'origine, ce décret a été adopté en vue d'établir la liste des communes dans lesquelles, en raison d'une tension sur le marché du logement, une taxe sur les logements vacants peut être instaurée. Quel est l'avis de la commission ? Favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Par cet amendement, au-delà de la régulation de l'activité dont il est question, et afin de ne pas encourager la soustraction de logements du marché locatif traditionnel, nous voulons poser la question du modèle même de ces plateformes, qui, sous couvert de souplesse, échappent totalement à l'impôt sur le territoire national. En effet, les maisons mères sont le plus souvent dans des pays que l'on peut qualifier de paradis fiscaux. Nous souhaitons que le Gouvernement place la lutte contre l'évasion fiscale comme une priorité absolue,

par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme

du chiffre d'affaires, mais des commissionnements opérés par la plateforme sur les transactions dont l'objet est un local situé en France. Cette taxe serait affectée au Fonds national des aides à la pierre, afin d'encourager la construction de logements abordables. Il s'agit symboliquement de faire contribuer à l'effort de construction les plateformes dont l'activité a trop longtemps induit le changement de destination de logements d'habitation en logements touristiques. Alors que l'instauration d'une telle taxe à l'échelon européen est en discussion, il serait pertinent que notre pays, sur ce combat, se place en premier de cordée.

L'équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, notamment la possibilité de recourir librement à la location saisonnière. location saisonnière. Cet amendement a donc pour objet de formaliser un régime dérogatoire à l'endroit des résidences universitaires, afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés

très temporairement de louer une chambre pour leurs activités. Pour ma part, je considère que c'est bien plus utile, en tout cas beaucoup plus encadré que le bail mobilité,

disposent de ressources largement inférieures au plafond d'accès au logement social et même, bien souvent, aux 60 %, niveau retenu pour l'attribution d'un PLAI.

000 à 5 000 logements mis sur le « marché « en flux annuel » -, singulièrement dans les secteurs locatifs nettement marqués par les désordres du marché, pose problème. Ces logiques de segmentation de l'offre de logement ont encouragé les inégalités et ségrégations spatiales, dont souffre notre pays et que nous cessons, depuis, de tenter de juguler. Cet article semble donc se fixer un objectif de « fluidification » du marché du logement, en proposant aux aspirants locataires une étape supplémentaire dans le parcours résidentiel, une étape située quelque part entre le loyer HLM. Cette réponse au « chaînon manquant » du déterminisme social de l'occupation locative ne nous paraît pas la meilleure. la meilleure. En effet, réaliser des logements, fussent-ils intermédiaires, dans des zones tendues appelle la réunion d'un certain nombre de critères, dont le moindre n'est pas de mobiliser un terrain d'assise pour l'immeuble ou les immeubles à construire. Sur un plan foncier et financier, le logement intermédiaire, grande spécialité de la Société nationale immobilière, n'est qu'une réponse imparfaite, notamment quand elle concerne des zones où les disponibilités foncières sont, par nature, assez rares et chères.

vaut également pour les villes et quartiers qui, de manière générale, ont sans doute un grand poids économique et politique, mais abritent aussi tant bien que mal une population souvent modeste et mal logée. La régulation du secteur locatif privé, qui reste à mettre en oeuvre, est plus pertinente que la généralisation de la production de PLI. Cela ne fait pas un pli ! Quel est l'avis de

à la constitution, dans tous les territoires tendus ciblés, d'une étape du parcours résidentiel, étape à ce stade souvent absente, entre le parc social et le parc privé. Cette mesure a pour objectif de permettre la fluidité des parcours

pour objet de rendre ce mécanisme plus attractif pour les investisseurs, en prévoyant que la pleine propriété, dans la limite maximale de 50 % des logements, peut être reconstituée au bout de douze années, au lieu de quinze. Cette réduction de la durée d'usufruit locatif est limitée au seul logement intermédiaire : la durée minimale de quinze années pour la part de logements en exploitation locative sociale reste sanctuarisée.

que j'ai cosigné. Il a été directement inspiré par ce qui se passe actuellement dans son département de la Gironde et touche une problématique majeure qui ne fait que se renforcer année après année. Le manque croissant de main-d'oeuvre saisonnière française, en viticulture notamment, déstabilise tout un territoire. En l'absence de candidatures issues du cru, les exploitations n'ont d'autre choix que de recourir à des travailleurs européens, qui arrivent dans le Médoc, ou encore dans le Libournais, dans des conditions qui ne sont acceptables par personne. Face à cette situation, les élus locaux sont impuissants et voient des personnes loger pendant plusieurs semaines dans des toiles de tente, au beau milieu de la campagne, sans eau ni électricité, ou encore des familles entières qui dorment dans leur voiture, juste devant la mairie du village. Cette situation est inacceptable. C'est une question de dignité humaine. Au-delà des actions à plus long terme en matière de formation, les élus locaux ont besoin que l'État endosse ses responsabilités et mette tout le monde autour de la table, et cela rapidement. L'adoption de cet amendement permettrait justement aux maires ou aux présidents des communautés de communes qui seraient concernés

En créant l'article 52 , la commission des affaires économiques du Sénat a souhaité modifier les dispositions législatives en vigueur afférentes aux modalités d'élaboration de la Convention relative au logement des travailleurs saisonniers devant être conclue dans les communes où les intercommunalités dites « de tourisme en faisant porter sur l'État la responsabilité de produire le diagnostic des besoins en logements, en lieu et place des communes ou des EPCI. Cette mesure va à l'encontre du processus consacrant les collectivités, tout particulièrement l'échelon intercommunal, comme l'échelon pertinent pour définir et mettre en oeuvre des politiques du logement et de l'habitat adaptées aux réalités locales. ailleurs, les intercommunalités communes concernées disposent de ressources et d'outils existants pour la réalisation de ce diagnostic, tels que les programmes locaux de l'habitat, les dispositifs d'observation ou encore le plan départemental du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées. Pour ces raisons, le Gouvernement n'était pas favorable à la proposition visant à faire porter la responsabilité du diagnostic et de l'élaboration de la Convention relative au logement des travailleurs saisonniers sur l'État, dans le cadre de la

Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d'économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d'Action Logement. Les sociétés d'économie mixte non agréées, ne gérant pas de logements sociaux, mais construisant des logements intermédiaires, ne peuvent cependant pas bénéficier de taux réduit de TVA pour la construction de logements locatifs même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements. Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d'économie mixte ne gérant pas de logements sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, afin de favoriser la production de logements intermédiaires.

telle uniformisation ne prend pas en compte la réalité du marché locatif et la diversité des situations locatives. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 53 . Quel est l'avis de la commission ? L'objet L'objet de cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a estimé que les limitations au droit de délivrer congé par le bailleur, dont la mise en oeuvre est pour le moins complexe, ne participent pas, de fait, à la fluidité du marché des biens occupés par des locataires. Peu de temps après avoir acquis un bien loué, l'acquéreur peut avoir besoin de vendre ou de reprendre le logement, en dehors de toute considération spéculative, à la suite d'un divorce, d'une mutation, d'une perte d'emploi

pour les baux d'habitation est de trois mois, sauf dans certaines zones dites tendues et pour certains motifs, que ceux-ci soient liés à l'emploi, à la santé, aux ressources, à l'attribution d'un logement social. Dans ces cas, le préavis est d'un mois. La commission a souhaité uniformiser les délais

et avoir des conséquences financières relativement importantes pour le locataire. Dès lors, il nous paraît tout à fait opportun de rétablir non

qui se voient attribuer un logement social. Si, dans le premier cas, la question peut effectivement se poser, dans le second, le délai de deux mois est inutilement long. En effet, le locataire concerné paiera un mois supplémentaire de loyer au prix du marché et, dans l'attente, le bailleur social risque de se retrouver avec un logement vacant pendant cette durée. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le délai de préavis à un mois pour le locataire amené à entrer dans le parc social. Quel est l'avis de la commission ? et ce sur l'ensemble du territoire. Sont néanmoins maintenues les exceptions abaissant ce délai à un mois pour les situations concernant l'état de santé du locataire et la situation économique difficile qu'il est susceptible de rencontrer. Il s'agit ainsi d'harmoniser et de simplifier, pour le locataire et le bailleur, les délais applicables.

par la loi ALUR a jeté un doute quant au maintien de cette prohibition. En effet, certains bailleurs arguent qu'ils n'encaissent pas les sommes d'argent en question, puisqu'elles sont déposées auprès d'un établissement tiers.

des établissements bancaires en ligne promouvant ainsi ce dispositif auprès des bailleurs. Elles précisent, par ailleurs, que les frais de gestion du compte sont à la charge du locataire. Dans les zones tendues, certains locataires sont contraints de se plier à ce type d'exigences. Aussi proposons-nous, par cet amendement, de reprendre la rédaction de la loi du 6 juillet 1989, avant sa modification par la loi ALUR, et d'étendre une telle interdiction aux locations meublées.

n'a toujours pas connu ne serait-ce que le début d'une mise en place ; elle a été remplacée par le dispositif VISALE, bien moins ambitieux et absolument pas universel. Comment se fait-il qu'un dispositif voté par les représentants du peuple puisse passer à la trappe sans bruit ni débat

À l'inverse des dispositifs prévus dans ce texte, qui précarisent les locataires, nous considérons qu'il convient de sécuriser les parcours résidentiels. Quel est l'avis de la commission ? Chacun l'aura

l'amendement qui nous est proposé pour engager le lancement opérationnel de la garantie universelle des loyers au 1 janvier 2019. Après concertation avec l'excellent secrétaire d'État,

Dallier, pour explication de vote. Je voudrais remercier nos collègues du groupe CRCE d'avoir, au sixième jour de débat, à minuit et quart, actionné la machine à remonter le temps, pour nous ramener quasiment cinq années en arrière, sur un sujet qui nous avait très longuement occupés sur toutes ces travées

L'article 53 C vise à autoriser l'insertion d'une clause pénale au sein du contrat de location, c'est-à-dire la possibilité, pour le bailleur, de prévoir une sanction en cas d'infraction à une partie des clauses du contrat de location ou du règlement intérieur à l'immeuble. Principalement, le bailleur pourra désormais prévoir, dans le contrat de location, des frais de retard en cas de non-paiement du loyer en temps et en heure. Si cet article vise à permettre aux propriétaires de dissuader les locataires de mauvaise foi qui payent leur loyer en retard, les raisons de ce retard ne pourront être prises en compte par les bailleurs souhaitant intégrer cette clause au contrat. Ainsi, lorsque le locataire est de bonne foi et que la situation est indépendante de sa volonté, des pénalités de retard pourront s'appliquer. Dans la mesure où les locataires qui ne respectent pas le délai pour payer leur loyer sont, pour l'écrasante majorité d'entre eux, en situation de surendettement, en proie à de fortes variations de salaires, comme c'est le cas des salariés de start-up, ou à des difficultés financières, laisser les bailleurs leur imposer des sanctions de leur propre chef n'aurait pour effet que de précariser d'autant plus les ménages les plus fragiles et les mal-logés, qui parfois doivent choisir entre se soigner, nourrir les enfants et payer le loyer. De plus, dans le contexte actuel, où le rapport de force sur le marché de l'immobilier est très défavorable au locataire, ce qui se traduit, notamment, par la cherté des loyers et des difficultés d'accès au logement, laisser la possibilité aux bailleurs de se faire justice eux-mêmes n'aurait pour effet que d'accroître

Il a beaucoup été question de l'équilibre entre bailleurs et locataires. Il vient d'être rappelé la situation des locataires, dans cette période de tension, avec un manque réel de logements à disposition.